J'informe le Sénat que la commission mixte paritaire chargée d'élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi portant création d'une taxe sur les services numériques et modification de la trajectoire de baisse de l'impôt sur les sociétés est parvenue à l'adoption d'un texte commun. L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée,

suscite d'ailleurs des mouvements de protestation inédits au sein du monde sportif, celui-ci n'étant pas habitué à se manifester de la sorte. C'est dire si l'heure est grave.

on brise toute la dynamique sportive et on court le risque d'un déclassement dans les prochaines années. Le sport doit être considéré non pas comme la variable d'ajustement budgétaire de notre pays, mais comme un investissement d'avenir. Il sert la cohésion sociale, la cohésion des territoires, l'entraide, la santé, le savoir et la connaissance. Arrêtons ce massacre, monsieur le secrétaire

aux fédérations sportives, que permet l'alinéa 11 de ce projet de loi. Les CTS occupent une place unique dans l'organisation du sport français et ont contribué à faire de la France l'un des pays qui ont le plus développé des politiques de sport de haut niveau et de sport pour tous. Ils sont au coeur de notre modèle sportif, qui s'est construit à partir des années soixante autour des structures associatives - les fédérations sportives agréées - et du ministère des sports, chargé d'apporter une expertise sous la forme de la mise à disposition de personnels qualifiés. Le rôle joué par les CTS est d'une importance d'autant plus capitale que la France s'apprête à participer aux jeux Olympiques et Paralympiques de Tokyo en 2020 et à organiser ceux de Paris en 2024. Ces échéances appellent la mobilisation de tous. Or celle-ci est menacée par la volonté du Gouvernement de transférer coûte que coûte les CTS aux fédérations sportives déléguées. Par ailleurs, ma collègue l'a dit, les petites fédérations sont particulièrement menacées par le détachement automatique, car, faute de moyens financiers, elles auront des difficultés à conserver les CTS qu'elles emploient et feront face à une situation de désorganisation totale. Aussi la prégnance des CTS au sein du système sportif français rend-elle inconcevable un transfert automatique qui n'a fait l'objet, à ce jour, d'aucune concertation avec les professionnels concernés et dont la possible compensation financière est loin d'être assurée.

ce qui laisse du temps à Mme la ministre des sports pour entamer le dialogue. Une concertation avec les représentants des CTS, des fédérations sportives et des collectivités locales, voire avec la nouvelle agence du sport, sur l'avenir de ces experts du sport afin de ne pas affaiblir les performances des athlètes français aux prochains jeux Olympiques et Paralympiques, singulièrement aux jeux de Paris en 2024, et de ne pas obérer la pérennité des plus petites fédérations.

Sa rédaction actuelle prévoit la possibilité, pour le fonctionnaire, de demander à mettre fin à son détachement. Cette demande peut être faite à tout moment, donc dès le prononcé de la décision de détachement. Par conséquent, il ne nous paraît pas nécessaire

Par sécurité, notre collègue Michel Savin, nommé rapporteur d'une mission d'information sur l'avenir des conseillers techniques et sportifs, ainsi que notre collègue Patrick Kanner proposent toutefois d'exclure la possibilité de détacher d'office les CTS actuellement en fonction auprès des fédérations sportives. Il nous semble effectivement nécessaire d'attendre les conclusions de la concertation engagée avant de prendre toute décision concernant l'avenir des CTS. La commission est donc favorable aux amendements identiques n 2 rectifié et 169

J'ai expliqué en quatre points en quoi ce dispositif était plus protecteur que le détachement volontaire, notamment en termes de salaire, de déroulement de carrière, de possibilité de retour dans l'emploi public avant terme et d'accompagnement, uniquement pour ceux qui le souhaitent, vers le secteur privé.

Nous recherchons d'autres objectifs. Je pense notamment aux conditions dans lesquelles nous pouvons déployer les maisons de services au public sur le territoire. la ministre des sports, vous l'avez dit à plusieurs reprises, s'est engagée au banc et je l'ai fait, au nom du Gouvernement, à l'occasion de l'examen de ce texte à l'Assemblée nationale, à ne pas utiliser

pour exiger que les CTS demeurent des agents de l'État en situation de mener des politiques publiques du sport. Nous regrettons que le Gouvernement, dans cette affaire,

nous sommes en pleine Coupe du monde de football féminin, à un an des jeux Olympiques de Tokyo, préparatoires de ceux de 2024, à trois ans de la Coupe du monde de rugby, qui aura lieu en France,

un climat anxiogène dans le monde du sport en supprimant des dispositifs qui fonctionnaient bien, comme le Centre national pour le développement du sport, en diminuant les moyens accordés au secteur associatif,

Si tous ces faisceaux de présomption ne vous alertent pas sur la grande inquiétude du monde sportif français, vous devenez aveugle et sourd

Marie. Cet amendement de repli tend à permettre aux fonctionnaires détachés d'office en cas d'externalisation de demander la fin de leur détachement pour pouvoir réintégrer leur corps ou leur cadre d'emploi d'origine. Actuellement, l'article 28 prévoit seulement que le fonctionnaire pourra demander qu'il soit mis fin à son détachement pour occuper un emploi au sein d'une des administrations mentionnées à l'article 2 du statut général. Cela ne lui garantit aucunement de retrouver son corps ou cadre d'origine.

au sein de la fonction publique. Le retour dans le corps ou le cadre d'origine de fonctionnaires dont les missions ont été transférées pourrait dans certains cas se révéler complexe à gérer. Surtout, les dispositions en vigueur offrent plus de possibilités aux fonctionnaires concernés, en leur permettant notamment d'intégrer un autre versant de la fonction publique que celui

L'article 28 comporte l'une des mesures les plus importantes et les plus polémiques du projet de loi. Il permet le détachement d'office des agents dont le service est externalisé. En effet, comme cela a été rappelé, les dispositions actuelles relatives au détachement permettent à l'argent de s'y opposer, ce qui complique considérablement les recours à l'externalisation. Les manifestations des gilets jaunes et le grand débat national ont une nouvelle fois mis en lumière l'insatisfaction de nos concitoyens quant à la qualité des services publics rendus au regard du niveau des prélèvements opérés. Cette insatisfaction doit mieux être prise en compte et se traduire par une réflexion globale sur le service public. Faut-il plutôt recentrer l'action des agents publics sur les missions régaliennes régaliennes ou adopter une démarche de recentrage guidée par l'analyse des efficiences relatives entre le secteur public et des services privés, comme le suggère le rapport Webhelp remis à Gérald Darmanin au mois de mars dernier ? Cette réflexion est absolument nécessaire. Dans plusieurs cas, on peut s'apercevoir que l'externalisation n'est pas la panacée. La multiplication des partenariats public-privé est désormais dans le viseur des observateurs des comptes publics et occupe nos magistrats financiers. Faute de vigilance ou de compétences de la part des décideurs publics, ces partenariats peuvent se révéler désastreux pour les deniers publics. préconise d'ailleurs des changements majeurs des dispositions relatives à la commande publique : l'introduction d'« une procédure d'évaluation obligatoire » ; « une approche partenariale de l'externalisation davantage tournée vers la performance » ; « le renforcement du suivi et la transparence de la gestion des services publics ». Ces dispositions ne sont pas abordées par le projet de loi, qui se borne à faire sauter l'une des plus grosses entraves à la décision d'externaliser.

est devenue une réalité dans la carrière de très nombreux fonctionnaires territoriaux occupant des emplois de direction. Cette procédure, qui présentait à ses débuts un caractère exceptionnel, est devenue relativement fréquente. Elle est aussi très souvent perçue comme une simple possibilité de mettre fin à la relation existante entre l'autorité de la collectivité locale et le directeur général. les professionnels qui accompagnent les agents en procédure de fin de détachement s'emploient désormais, et c'est positif, à favoriser la mobilité, et non à s'enfermer dans des logiques de contentieux inutiles.

pourrait s'appliquer comme une période de préavis préalable à l'enclenchement de la procédure permettant d'engager les démarches en vue d'une mobilité. Un protocole négocié pourrait organiser cette période de transition. Il pourrait également être proposé la création d'un nouveau délai minimal d'un mois entre l'entretien préalable et l'information faite à l'assemblée délibérante. Je le précise, cet

Les fonctionnaires détachés sur un emploi fonctionnel d'une collectivité territoriale bénéficient de certaines garanties au terme de leur détachement. Il ne peut être mis fin à leurs fonctions qu'après un délai de six mois suivant soit leur nomination dans l'emploi, soit la désignation de l'autorité territoriale. La fin des fonctions est précédée d'un entretien entre l'autorité territoriale et les intéressés. Elle ne prend effet que le premier jour du troisième mois suivant la date à laquelle l'assemblée délibérante en a été informée. Cet amendement tend à mieux tirer parti du délai de six mois qui doit s'écouler entre l'élection d'un nouvel exécutif et la cessation des fonctions du fonctionnaire. Ce laps de temps serait transformé en un délai de préavis, et l'agent serait autorisé pendant cette période à rechercher une nouvelle affectation « en

J'y suis donc plutôt favorable. Néanmoins, ainsi rédigé, un tel dispositif empêcherait un employeur public territorial en cours de mandat de mettre fin aux fonctions des personnes intéressées avant six mois, et même dix mois, puisqu'il faudrait y ajouter quatre mois de procédure liée à l'entretien préalable et à l'information de l'organe délibérant. Cela ne me paraît pas opportun. Je vous soumets donc un sous-amendement, mes chers collègues, visant à préciser la rédaction proposée, à maintenir les délais actuels tout en permettant qu'ils soient employés à bon escient pour faciliter la mobilité de l'agent et à étendre les dispositions proposées aux fonctionnaires détachés en qualité de directeur départemental ou directeur départemental adjoint des services d'incendie et de secours.

En effet, cet article s'attaque à la garantie d'emploi des fonctionnaires territoriaux. Or cette garantie est, rappelons-le, le corollaire d'un traitement souvent bien moins intéressant que dans le privé.

statutaires relatives à la fonction publique territoriale, le fonctionnaire territorial dont l'emploi est supprimé est placé pendant un an en position de surnombre dans son administration d'origine, puis pris en charge par le Centre national de la fonction publique pour les emplois fonctionnels, ou par les centres de gestion, pour les autres emplois. Pendant cette prise en charge, l'agent est placé sous l'autorité du CNFPT ou du centre de gestion. de gestion. Il est soumis « à tous les droits et obligations attachés à sa qualité de fonctionnaire » et tenu de suivre « toutes les actions d'orientation, de formation et d'évaluation destinées à favoriser son reclassement

Dans un contexte de concurrence accrue entre fonctionnaires et contractuels du fait d'un renforcement des possibilités de recrutement sur contrat, une telle disposition constituera une double peine pour les fonctionnaires dont

que ces quelque 400 fonctionnaires ne feraient pas les efforts nécessaires pour retrouver un poste. C'est particulièrement condamnable de penser cela. La plupart de ces agents souhaiteraient se repositionner, mais éprouvent des difficultés pour le faire. Il nous paraît totalement incorrect de devoir les licencier au bout de cinq ans. Nous voulons donc la suppression de cet article.

est l'avis du Gouvernement ? Le Gouvernement partage l'objectif de la commission des lois de limiter dans le temps la prise en charge des fonctionnaires momentanément privés d'emploi.

précisions sur la durée de prise en charge, que nous proposons de porter de cinq ans à dix ans. En contrepartie, nous prévoyons des mesures incitatives pour que les centres de gestion puissent engager plus d'actions en matière d'accompagnement, de réinsertion et de reclassement des agents concernés.

ensemble. Cet amendement de compromis vise à durcir le dispositif de dégressivité de la rémunération des FMPE et à préciser les cas de licenciement des FMPE, notamment lorsqu'ils ne seront plus rémunérés.

le fonctionnaire détaché, qui ne peut retrouver un emploi dans sa collectivité d'origine, est en principe régi par les dispositions relatives aux fonctionnaires momentanément privés d'emploi.

En outre, les fonctionnaires à temps plein ou à temps non complet qui sont pris en charge se voient souvent proposer un reclassement à temps non complet, donc en deçà de leur durée d'emploi prise en charge. Aussi, il conviendrait selon nous d'aménager les dispositions permettant leur reclassement dans un emploi à temps non complet. Le reliquat d'heures dans le cadre de la prise en charge serait naturellement maintenu par le centre de gestion ou par le CNFPT. Quel est l'avis de

avec des variations entre les versants. L'écart était de 20,6 % dans la fonction publique hospitalière, de 14,3 % dans la fonction publique de l'État et de 9,1 % dans la fonction publique territoriale.

publics, la réalisation d'un plan d'action relatif à l'égalité réelle. En cas de non-respect de cette obligation, une sanction financière équivalant à 1 % de la rémunération brute annuelle globale du personnel pourra être appliquée.

malgré les dispositifs légaux mis en place depuis 2001 et surtout après 2012, ces inégalités salariales se résorbent très seulement. L'écart n'a été porté que de 13,1 % à 12,9 % entre 2015 et 2016, et 2016, et cette moyenne cache des réalités très variables d'un versant à un autre : dans la fonction publique hospitalière, où les femmes représentent 78 % des effectifs, l'inégalité salariale constatée est de 20,6 Dans la fonction publique de l'État, elle est de 14,3 %. De son côté, la fonction publique territoriale fait office de bon élève, avec le plus faible écart observé, 9,1 % : les employeurs locaux apparaissent donc plus vertueux que les autres employeurs publics.

supprimer la définition de cet état de situation comparée par un décret en Conseil d'État, dès lors que le fonctionnement actuel ne semble pas avoir présenté de dysfonctionnement de nature à le justifier : il faut éviter d'engorger la haute juridiction. Quel

: La parole est à Mme Éliane Assassi. Nous proposons de renforcer le dispositif de signalement par un dispositif d'accompagnement des victimes de violences sexistes et sexuelles. Pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles, les mesures prévues à l'article 29 se contente de créer une procédure de signalement, alors que les besoins sont particulièrement forts. Si l'étude d'impact ne fournit pas de données chiffrées quant aux violences sexuelles, elle évoque tout de même 98 sanctions disciplinaires prononcées contre des agents publics, en 2017, pour fautes graves relatives aux moeurs. Parmi celles-ci figure le harcèlement sexuel. Pour rappel, 80 % des femmes déclarent être victimes de sexisme au travail et 20 % de harcèlement sexuel. Dix viols ou tentatives de viol ont lieu chaque jour

du problème leur a été défavorable : elles ont été mutées, placardisées ou licenciées. Ce dispositif vise également à prendre en compte les situations de violences subies et repérées sur le lieu de travail, en prévoyant un accompagnement, une protection et un suivi de la victime. À l'image du bilan social annuel, un bilan

commission ? L'amendement n° 264 nous semble satisfait. Le dispositif de signalement vise à orienter la victime vers les autorités compétentes en matière d'accompagnement et de soutien. Il peut être utilisé par les témoins de violences sur le lieu de travail.

est à Mme Laurence Rossignol. Cet amendement vise à compléter le dispositif de lutte contre les violences sexuelles et sexistes dans l'entreprise, en l'occurrence dans les établissements de la fonction publique- les administrations, les collectivités -, en prévoyant la désignation d'un référent

penser qu'en l'absence d'un référent clairement identifié les victimes ne savent pas comment se faire entendre. Elles ignorent si elles vont prendre des risques

pour prévenir les causes et les situations de violences. De même, le référent doit être en mesure d'accompagner la victime dans ses démarches. Une telle fonction ne s'improvise pas. C'est pourquoi nous proposons d'instituer un droit d'alerte du référent, afin qu'il puisse déclencher immédiatement une enquête paritaire avec l'employeur, qu'un droit de recourir à un expert dans le domaine des violences sexuelles et sexistes pour l'aider dans sa mission. Enfin, pour mener à bien sa mission, le référent en matière de lutte contre les violences sexuelles et sexistes doit bénéficier

un dispositif qui a pour objet de recueillir les signalements des agents qui s'estiment victimes d'un acte de violence, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel ou d'agissements sexistes et de les orienter vers les autorités compétentes en matière d'accompagnement et de soutien des victimes et de traitement des faits signalés. » Je précise, évidemment, qu'il s'agit d'un dispositif mis en oeuvre en amont du dépôt de plainte proprement dit. dit. Ces deux amendements visent, selon des modalités différentes, à instituer des référents pour accompagner les victimes de violences sexuelles ou sexistes et suivre leur signalement.

effet tout en oeuvre avec l'équipe qui est la mienne pour faire en sorte que l'égalité et le refus des discriminations soient au coeur de toutes nos priorités. J'ai engagé des campagnes de testing anonyme sur les conditions de recrutement et les possibilités de discrimination fondées sur l'orientation sexuelle, l'identité de genre et les comportements sexistes

Nous veillons à ce que les membres des jurys soient tous sensibilisés à la question du refus des discriminations, qu'elles soient fondées sur l'identité ou l'orientation sexuelle, sur les origines ethniques, sur la confession religieuse, de manière que l'égalité soit partout présente. Je veille aussi à ce que les acteurs de la lutte contre les discriminations sexistes ou sexuelles, ou fondées sur l'orientation ou l'identité de genre soient accompagnés par mes services. J'ai mené les négociations autour du protocole d'accord sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes avec cet objectif. Nous avons renforcé les dispositions en matière d'accès aux responsabilités

que les avancées proposées dans les articles relatifs à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes soient validées et soutenues par l'intégralité des employeurs des trois versants

Un des engagements que j'ai pris devant les neuf organisations syndicales signataires ou non et l'ensemble des employeurs territoriaux était de veiller à la fidélité de la transposition dans la loi des dispositions contenues dans l'accord.

je reste aussi fidèle à mon engagement de transposition aussi conforme que possible de l'accord. Je note, pour la bonne information du Sénat, qu'en matière de plans de réduction des inégalités de salaires, notamment,

Pour autant, même si je vous souhaite une très longue vie ministérielle, je ne suis pas sûre que nous arrivions, pendant le temps où vous occuperez ce poste, à éradiquer les violences sexuelles.

l'ambition que doit avoir chaque titulaire de ce portefeuille en termes de durée et de capacité à atteindre l'égalité entre les femmes et les hommes. Je pense même que plusieurs de mes successeurs auront encore un peu de travail en la matière.

M. Didier Marie. L'article 29 prévoit notamment que les communes et établissements publics de coopération intercommunale de plus de 20 000 habitants devront élaborer et mettre en oeuvre un plan d'action pluriannuel en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. L'effectif de la population nous paraît avoir peu

personnelle, discriminations, actes de violence, harcèlement. C'est donc bien en référence aux agents et à leur effectif qu'il faut rendre ou non applicable ce dispositif. Cela nous paraîtrait plus pertinent.

de la commission ? L'article 29 crée une obligation d'élaborer un plan d'action pluriannuel pour l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, d'une durée maximale de trois ans, et de le mettre en oeuvre. S'agissant des communes et EPCI, cette obligation était initialement prévue à partir d'un seuil de 40 000 habitants dans l'accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la fonction publique du 30 novembre 2018, que M. le secrétaire d'État a évoqué. Ce seuil a été abaissé à 20 000 habitants lors de la discussion au sein du Conseil commun de la fonction publique, ce qui porterait à 2 100 le nombre de collectivités concernées, au lieu des 1 100 envisagées

Mme Laurence Cohen. Les obligations de l'article 29, nous l'avons souligné, sont largement insuffisantes pour atteindre l'égalité des droits et des rémunérations entre les femmes et les hommes dans la fonction publique. Le plan d'action pour réaliser l'égalité réelle peut être un outil pertinent

l'avis de la commission ? Le terme « traiter » me semble plus approprié que le terme « supprimer ». Il laisse de la souplesse aux employeurs publics pour apporter une réponse, éventuellement échelonnée dans le temps, aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes. La commission émet donc un avis

de ces inégalités et, nous l'espérons, du coût de ces réductions. Je rappelle que, le 8 mars dernier, nous avons présenté aux partenaires sociaux la méthodologie selon laquelle nous voulons construire ces indicateurs. Je crois pouvoir assurer que celle-ci a été approuvée par tous, considérant qu'elle était suffisamment complète pour donner une véritable vision et une réelle capacité de lecture des inégalités, et donc une meilleure capacité à les combattre. La parole est à Mme Laurence Cohen, pour explication de vote.

et qu'elle recelait même quelques dispositifs internes, pratiques, coutumes et habitudes qui y rendent la question de l'égalité professionnelle peut-être encore

la mesure des écarts de rémunération entre femmes et hommes. Il s'agirait ainsi de mettre à la charge des employeurs publics une nouvelle formalité administrative qui nous semble peu opérationnelle. En effet, cette information figurera dans le rapport social unique prévu à l'article 3 A, qui intégrera des indicateurs relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, et qui sera rendu public après débat devant les comités sociaux. L'avis est donc défavorable.

parole est à Mme Laurence Cohen. Nous demandons que soient garanties chaque année la continuité et la dynamique du plan institué par le présent article. Pour ce faire, nous proposons qu'un bilan annuel de la mise en oeuvre du plan soit prévu dans chaque rapport de situation comparée, intégré par cet article rapport social unique. Rappelons-nous que le rapport de situation comparée entre les hommes et les femmes dans les services et les établissements des trois versants de la fonction publique a été institué en 2012 par par la loi Sauvadet et qu'il est annuel, alors que le plan d'action est pensé sur une durée de trois années. Nous estimons qu'il est nécessaire de revenir chaque année sur les avancées réalisées en intégrant au rapport social unique un bilan de celui-ci. Je pense que nous pouvons partager cet objectif, mes chers collègues, monsieur le secrétaire d'État, car nous voyons

Le texte initial prévoyait la « possibilité » de sanctionner par une pénalité financière la non-élaboration du plan d'action, en renvoyant à un décret en Conseil d'État. Si le montant d'une pénalité peut dépendre d'un décret en Conseil d'État, son principe doit, lui, être fixé dans la loi. C'est pourquoi la commission a remplacé

certainement progressifs, de cette pénalité seront fixés par décret. Pour ce qui concerne les collectivités locales et les établissements hospitaliers, il y aura une forme de contrôle de légalité. L'État devra s'appliquer à lui-même la pénalité, ce qui n'est ni une rareté ni une nouveauté. En effet, concernant les obligations de nominations équilibrées, le le dispositif de pénalités financières est contrôlé par l'État pour lui-même. Je saisis cette occasion pour vous dire que, en 2019, pour la première fois, l'intégralité des employeurs publics des trois versants soumis à pénalité financière pour manquement à l'obligation de nominations équilibrées ont versé la contribution.

Nous sommes donc bien évidemment opposés à l'amendement du Gouvernement. Dire qu'il « peut » y avoir une pénalité financière, c'est laisser la porte ouverte à une forme d'arbitraire. En vertu de quels critères, entre deux employeurs ne respectant pas l'obligation d'élaborer un plan d'action,

Près des deux tiers des emplois de la fonction publique sont occupés par des femmes selon les données publiées par le ministère de l'action et des comptes publics. Un secteur largement féminisé, contrairement au secteur privé. Mais la présence des femmes s'amenuise à mesure que l'on grimpe dans la hiérarchie. Elles ne sont que 41 % à occuper un emploi d'encadrement supérieur et de direction. » La fonction publique est bien souvent novatrice dans la manière d'envisager le travail de ses agents elle occupe à plus d'un titre une place singulière dans le monde du travail. Nous nous devons en retour, mes chers collègues, de la doter d'outils solides pour l'avenir, afin de faire de l'égalité entre les femmes et les hommes une réalité. L'amendement

Ces amendements tendent à augmenter le montant maximal de la pénalité financière encourue en cas de non-respect de l'obligation d'élaborer un plan d'action pour assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Ce montant

La sanction prévue, équivalente à celle d'ores et déjà appliquée dans le secteur privé, semble suffisamment dissuasive. L'avis est donc défavorable.

M. Arnaud de Belenet. Il est désormais bien établi que le recours effectif à l'article 40 du code de procédure pénale par les fonctionnaires demeure peu conciliable avec les obligations statutaires diverses qui sont imposées aux agents publics. Et pour cause : le devoir de réserve, l'obéissance hiérarchique ou encore la loyauté sont autant de prescriptions de service qui acclimatent le fonctionnaire à une forme de retenue, parfois même au prix de quelques injonctions contradictoires.

il rappelle que tout fonctionnaire qui engage sur la base de soupçons raisonnables, et de bonne foi, la procédure prévue au second alinéa de l'article 40 du code de procédure pénale ne doit subir aucune sanction disciplinaire ou mesure discriminatoire. En second lieu, il précise que tout fonctionnaire qui acquiert dans l'exercice de ses fonctions la connaissance d'un crime ou d'un délit peut témoigner de tels faits auprès du référent déontologue. Quel est l'avis de la commission ? La

protège déjà contre d'éventuelles représailles les fonctionnaires ayant signalé aux autorités judiciaires des faits constitutifs d'un délit ou d'un crime. Par ailleurs, s'agissant de l'intervention du référent déontologue soit les faits relèvent de la déontologie, et il est déjà compétent- avec les notions de « dignité, impartialité, intégrité et probité », la déontologie appréhende de nombreux faits susceptibles d'être qualifiés de délits ou de crimes soit il s'agit de faits qui ne relèvent que du champ pénal et il ne me semble pas opportun d'ajouter de nouvelles compétences au référent déontologue, au risque de lui faire perdre sa spécificité. L'avis est défavorable. Quel est l'avis

M. Didier Marie. Cet amendement tend à compléter les critères de discrimination mentionnés à l'article 6 du statut général, de façon à aligner les régimes applicables au secteur privé et au secteur public, ce dernier ne pouvant être moins-disant que ce que prévoit le code du travail. à interdire toute discrimination fondée sur les caractéristiques génétiques, la particulière vulnérabilité résultant de la situation économique, le lieu de résidence ou de domiciliation bancaire, et sur la capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français. Il intègre, bien entendu, le critère de discrimination en raison de l'état de grossesse adopté à l'Assemblée nationale. Enfin, sur recommandation du Défenseur des droits, et toujours par cohérence avec le code du travail, l'amendement fait référence à la loi du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, qui définit les différentes formes de discrimination- discrimination directe et indirecte, harcèlement à caractère discriminatoire, mesures de rétorsion -et envisage les différentes manifestations de la discrimination par une décision, un agissement.

pose le principe de l'interdiction des discriminations fondées sur les opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, l'origine, l'âge, le handicap. Cette liste est augmentée au fil des lois et devient de plus en plus précise, ce qui risque de priver le juge ou le pouvoir disciplinaire de toute marge d'interprétation. Or toutes les situations rencontrées ne peuvent pas être couvertes explicitement par la loi.

un dispositif pour les emplois de direction. Nous vous proposons de l'élargir aux emplois de sous-direction, de chef de bureau, sous-directeur et équivalents, justement, pour

commission ? L'article 30 du projet de loi vise à étendre l'obligation de nominations équilibrées dans les emplois supérieurs et de direction de la fonction publique en élargissant le champ des emplois et des administrations concernées. Les auteurs de l'amendement souhaitent aller plus loin en faisant entrer dans le champ du dispositif des emplois de sous-direction, chef de bureau, sous-directeur et équivalents. S'agissant des sous-directeurs, il me semble que l'amendement est pour partie satisfait. En effet, le décret du 30 avril 2012 vise expressément les sous-directeurs des administrations de l'État et de ses établissements publics parmi les emplois de type 2. Par ailleurs, nous pensons que l'obligation de nominations équilibrées est déjà suffisamment contraignante pour les employeurs Si l'obligation ne vise que les emplois d'encadrement supérieur, elle a un effet positif plus général sur la carrière des femmes, puisqu'elle suppose que les employeurs disposent en amont d'un vivier suffisant de femmes promouvables. L'avis est donc défavorable. Quel est l'avis du Gouvernement ?

une répartition équilibrée, ou en tout cas conforme, entre les femmes et les hommes des promotions et des avancements au choix, en conformité avec les corps et les cadres d'emplois concernés.

S'agissant des postes de chef de bureau, ceux-ci ne relèvent d'aucun texte réglementaire en termes de statut d'emploi particulier, contrairement aux autres emplois listés, et recouvrent des situations très diverses selon les administrations, ce qui rend difficile l'adoption des

diversifier le vivier est de faire en sorte que l'accès à la promotion et à l'avancement soit plus représentatif de la répartition femmes-hommes. La loi le prévoit, et c'est une avancée que je ne me lasse pas de souligner. La parole est

les effets. Si la loi de 1983 et le décret de 2012 atteignaient réellement leur objectif et satisfaisaient l'amendement que nous proposons,

C'est pourquoi il est proposé d'y adjoindre les emplois de responsabilité supérieure des juridictions judiciaires, administratives- Conseil d'État, cours administratives d'appel, tribunaux administratifs -et financières- Cour des comptes et chambres régionales et territoriales des comptes. Cet amendement vise à intégrer les emplois de responsabilité supérieure des juridictions judiciaires, administratives et financières dans le champ d'application de l'obligation de nominations équilibrées. L'intention est bonne, mais il nous semble que ces nominations doivent faire l'objet de procédures spécifiques, en particulier les nominations des magistrats judiciaires qui doivent recueillir l'avis du Conseil supérieur de la magistrature, le CSM, voire dans certains cas être directement proposées par le CSM. Le dispositif proposé ne nous semblant pas opérant

au principe d'indépendance de la magistrature et aux procédures de nominations soumises à avis ou à proposition du CSM. Les participants à la discussion autour de l'accord du 30 novembre dernier ont acté cette difficulté. L'action 2.3 du protocole d'accord prévoit que le travail doit continuer sur cette question, pour aboutir- effectivement avec un décalage dans le temps -sur ces questions d'emplois supérieurs dans les juridictions.

Il est défendu. Ces nominations ont été exclues afin de ne pas pénaliser les personnes déjà nommées sur des emplois de direction. Le mécanisme opère ainsi une conciliation entre l'objectif de rendre effectif l'égal accès aux emplois de direction entre les femmes et les hommes, et la préservation du déroulement de carrière des personnes en place. Cet équilibre doit être maintenu. L'avis est donc défavorable.

à M. Didier Marie. Cet amendement prévoit une montée en charge de la proportion minimale de personnes de chaque sexe devant être « primo-nommées » dans les emplois de direction de la fonction publique. Sous le précédent quinquennat, cette proportion est passée de 20 % en 2013 à 40 % en 2017, produisant des effets très positifs en termes de féminisation des emplois de direction. Si le Gouvernement proclame l'égalité entre les femmes et les hommes grande cause du quinquennat, il ne prévoit pourtant aucune nouvelle trajectoire de montée en charge de ce dispositif. Pourtant, le taux de 40 % est seulement une étape sur le chemin de l'égalité professionnelle, et pas une fin en soi. C'est la raison pour laquelle nous proposons d'établir à au moins 45 % cette proportion en 2022, puis à au moins 50 % en 2025.

de la commission ? L'amendement n° 174 rectifié vise à augmenter la proportion minimale de personnes de chaque sexe devant faire l'objet d'une primo-nomination. La proportion est actuellement de 40 %. Les auteurs souhaitent l'augmenter à 45 % en 2022, puis 50 % en 2025. L'amendement n° 175 rectifié est un amendement de repli qui fixe ce taux à 45 % en 2022. Nous pensons qu'il faut garder le taux de 40 % qui offre de la souplesse aux employeurs publics, surtout dans le versant territorial où parfois peu de nominations sont concernées. Je fais observer, comme je l'avais fait d'ailleurs en commission, que cet amendement peut se retourner contre les femmes elles-mêmes. En effet, dans un certain nombre d'administrations où elles sont d'ores et déjà majoritaires,

Marie. Il s'agit de supprimer l'alinéa 9 de l'article 30. La dérogation prévue à cet alinéa aura des effets pervers : la dispense de 40 % de primo-nominations de personnes de chaque sexe, au prétexte qu'il existe déjà ce ratio de 40 % en « stock », a pour effet de réduire mécaniquement ce stock. De plus, les femmes pourraient être concentrées sur la partie « basse » de l'enveloppe d'emplois, par exemple les postes de sous-directrices, tandis que les emplois plus élevés- directeurs généraux, secrétaires généraux -pourraient être occupés par des hommes, tout de même un affichage global de 40 %. En outre, l'absence de primo-nominations peut avoir ultérieurement un effet à la baisse, dès lors qu'une première nomination est un palier nécessaire dans les ministères où les carrières sont très linéaires. La dispense peut donc avoir un impact sur les parcours qualifiants, et faire disparaître des cohortes les femmes qui n'ont pas été nommées à des postes de direction et ne pourront pas candidater aux plus hauts postes par la suite. C'est dix ans plus tard que s'observeront les effets pervers et d'éviction de cette dérogation. Il importe donc de supprimer cette disposition.

Si l'on ne peut supprimer la dispense de sanction, cet élément de souplesse doit être encadré, sous peine de voir la trajectoire positive s'inverser. Il ne s'agirait pas qu'un employeur public, au motif que les effectifs globaux remplissent les obligations légales, renonce plusieurs années de suite à son obligation annuelle relative aux primo-nominations. C'est la raison pour laquelle nous proposons de limiter dans le temps cette dispense de sanction pour prévoir qu'elle ne peut être mise en oeuvre deux années consécutives. Quel est l'avis de la commission ? L'amendement n° 358 vise à revenir sur

L'amendement n° 191 rectifié tend à supprimer la dispense de pénalités accordée aux employeurs ayant déjà atteint la proportion de 40 % de personnes de chaque sexe dans leur « stock » d'emplois de direction. Les signataires de cet amendement expriment la crainte de voir diminuer le « stock » de femmes nommées sur ces emplois de direction. Nous pensons qu'il faut responsabiliser les employeurs publics : c'est à eux de veiller à maintenir cet équilibre de 40 % en procédant aux nominations adéquates. À défaut, ils retomberaient sous le coup d'une pénalité financière. L'avis est donc également défavorable. Enfin, sur l'amendement n° 176 rectifié qui prévoit d'encadrer cette même dispense pour la limiter dans le temps, même avis que précédemment, pour les mêmes raisons.

mais qu'elle augmente chaque année. C'est ce qui avait déjà été fait entre 2013 et 2017, puisqu'elle était de 30 000 euros en 2013, contre 90 000 euros en 2017. L'intérêt d'une telle mesure est d'éviter que les administrations n'intègrent dans leurs

L'amendement n° 187 rectifié vise à fixer dans la loi le montant de la pénalité due en cas de non-respect de l'obligation de nominations équilibrées et à l'augmenter. La contribution financière due est égale au nombre de nominations manquantes dans le périmètre considéré, multiplié par un montant fixé par décret qui est actuellement de 90 000 euros.

que les pénalités versées au budget général seront aussi utilisées pour des actions en matière d'égalité entre les femmes et les hommes. Nous avons créé un fonds pour l'égalité femmes-hommes par arrêté. Nous avons lancé un premier appel à projets, dont les résultats ont été rendus la semaine dernière. Nous pouvons, par la mobilisation de fonds équivalents aux pénalités, accompagner 42 projets sur l'égalité entre les femmes et les hommes dans la fonction publique. Nous avons donc préféré élargir l'assiette avec un prélèvement à niveau constant plutôt que de renforcer le taux, comme vous le proposez, madame la sénatrice. Ce sont les raisons pour lesquelles l'avis est défavorable,